Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, mesdames, messieurs les sénateurs,

je voudrais simplement rappeler d'où vient notre pays en termes de finances publiques et de situation économique. Nos finances publiques, c'est l'histoire d'une lente dégradation depuis quinze

elle est passée de 52 % à 55 % de notre richesse nationale. Trois, c'est également l'augmentation des taxes et des impôts : sur dix ans, ils

que nous réduisions par conséquent la dette et que nous puissions, au bout du compte, baisser les impôts et les taxes des Français. Je crois inutile d'insister sur la situation politique et sociale actuelle.

maintenant sortis de la procédure pour déficit public excessif, dans laquelle nous étions depuis dix ans. C'est un fait ! La réalité, c'est que nous sommes la première majorité, depuis dix ans, à passer sous les 3 % de déficit public. C'est un fait

qui est la nôtre et la réduction des charges qui pèsent sur la compétitivité-coût de notre industrie. Nous devons aussi continuer à innover et à investir pour la recherche, pour l'innovation, pour l'innovation de rupture dans notre pays.

une centaine d'entreprises qui ferment chaque année, des territoires comme le mien, l'Eure, où des vallées industrielles entières disparaissent : c'est le fruit de choix de politique économique qui n'ont pas été les bons. Tout ce que nous faisons actuellement- restauration des marges des entreprises, fiscalité qui permet de diminuer le coût du capital et donc d'investir, création d'un fonds pour l'innovation de rupture financé par la vente d'actifs de l'État dans des entreprises qui ne sont pas nécessairement stratégiques -tout cela doit permettre de redresser notre industrie. Ces choix de restauration des finances publiques et de relance de l'activité économique sont d'autant plus importants dans l'environnement que vous connaissez, qui est instable et menaçant pour notre économie.

La suppression du forfait social de 20 % sur l'intéressement pour toutes les entreprises de moins de 250 salariés, c'est plus de salaire net pour tous ceux qui travaillent et dont l'entreprise réussit. La suppression des cotisations sociales sur les heures supplémentaires à partir de 2019, ce sera aussi plus de salaire net pour ceux qui travaillent. Nous voulons que tous ceux qui travaillent,

Le suramortissement que nous vous proposons, conjugué à la baisse de l'impôt sur les sociétés, massive dès l'année prochaine, doit permettre à nos entreprises de se digitaliser et de réussir leur transition technologique. Le troisième choix que nous faisons- je sais qu'il fait débat aujourd'hui -, c'est celui de l'environnement.

notamment la convergence entre le diesel et l'essence, tout en accompagnant les Français dans cette transition écologique avec un crédit d'impôt spécifique et la prime à la conversion.

Nous allons également accompagner, à travers plusieurs mesures, les secteurs concernés par la hausse du tarif du gazole non routier, prévue à l'article 19 du projet de loi de finances. Des efforts sont aussi demandés aux entreprises.

J'entends certains de nos partenaires européens nous expliquer que la force de la zone euro ne tiendra qu'aux efforts nationaux produits par les États membres. Je reconnais bien volontiers que chaque État doit respecter les règles qu'il a librement et souverainement choisies. Il est essentiel, pour la cohésion de la zone, que ces règles soient respectées et que chacun se sente solidaire de leur respect, mais il est

Les choix que nous faisons aujourd'hui en matière de finances publiques visent à nous libérer de la contrainte de la dette et à nous redonner notre souveraineté financière. Ils nous permettent d'investir dans l'avenir de nos enfants et dans les ruptures technologiques, sur lesquelles la Chine et les États-Unis sont en train de prendre une avance que nous ne rattraperons pas, si nous n'y prenons pas garde.

Il n'est certainement pas encore assez élevé, mais je vous rappelle que nous n'avons pas connu trois années successives de croissance supérieure à 1,5 % depuis dix ans. Quelles étaient les hypothèses de déficit public, lorsque le Parlement a eu à connaître des chiffres du Gouvernement ? Respectivement, 2,8 % et 2,9 % du PIB en 2018 et en 2019. Et quelles sont les hypothèses retenues dans ce budget ? Pour 2018, 2,6 % et, pour 2019, 2,8 %, alors même, je l'ai dit, que nous avons intégré la dette de SNCF Réseau dans les comptes publics

La moindre des choses que nous devons au Parlement, c'est la vérité des comptes afin qu'ils correspondent effectivement aux projections et aux factures que paye notre pays ! Nous parviendrons à de tels résultats, en poursuivant la réduction de l'évolution de la dépense publique. Pour la première fois, de 0 % en volume en 2018, puis de 0,6 % en 2019, soit une progression bien inférieure aux moyennes constatées durant les trois dernières mandatures. Nous proposons ainsi l'évolution de la dépense publique la plus basse depuis quinze

Au cours des débats qui nous ont animés l'an passé et en ce début d'année, j'ai fréquemment insisté sur trois points de méthode, qui me semblent partagés par la grande majorité de cette assemblée plus de sincérité dans les comptes publics, plus de lisibilité dans la politique fiscale et moins de verticalité, notamment dans les relations entre l'État et les collectivités locales.

En ce qui concerne le troisième engagement que j'ai mentionné, j'ai le plaisir de vous indiquer la réussite de la contractualisation avec les collectivités locales les plus importantes. Je rappelle à cette occasion que, contrairement à ce que j'ai pu entendre ici ou là,

Nous confirmons les engagements présidentiels, notamment en faveur des ménages qui travaillent et des entreprises. Ainsi, l'année 2019 sera marquée par le plein effet sur les salaires de la suppression des cotisations chômage et maladie pour les salariés et les trois quarts des indépendants. Nous conjuguons cette mesure avec la désocialisation, un

de seuil supprimés et une meilleure répartition entre le capital et le travail. Je veux parler du forfait social ou encore de la participation. Nous aurons sans doute des débats autour de la fiscalité agricole, qui, si elle a fait pousser un certain nombre de sujets lors du PLFSS, est bénéfique

Nous aurons l'occasion d'évoquer les augmentations de crédits très importantes dans des domaines que le Gouvernement a choisis, avant tout dans le régalien : la défense, les forces de sécurité et de justice

que l'année dernière, ce qui est une bonne chose. C'est notamment grâce au Grand plan d'investissement qu'a mis en place le Gouvernement au début de l'année dernière. Nous avons fait le choix de l'environnement et des mobilités, comme l'a dit M. le ministre de l'économie et des finances. Nous prévoyons déjà

Le choix en faveur de l'avenir, c'est également le choix en faveur de l'éducation de nos enfants, qu'il s'agisse de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur, avec plus d'un milliard d'euros de crédits pour le monde éducatif. Il s'agit de la plus grande hausse en proportion qu'ont connue les ministères de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, ce dernier devant notamment accueillir 40 000 étudiants supplémentaires chaque année. C'est effectivement un sujet très important de discussion pour l'avenir de nos enfants. Les transformations de l'action publique sont nombreuses. J'évoquerai d'abord la décrue des effectifs de l'État et de ses opérateurs, avec une proposition de 4 200 suppressions de postes l'an prochain en net. Nous aurons l'occasion d'y revenir, notamment dans la trajectoire qui nous mène effectivement aux 50 000 suppressions de postes figurant dans le programme présidentiel. l'indispensable réflexion autour de l'offre audiovisuelle, avec le début de la réforme audiovisuelle publique, telle qu'elle a été annoncée par le Gouvernement l'année dernière. Il y a aussi la question, très importante évidemment, de la suppression des impôts qui vont avec la taxe d'habitation, ou l'accompagnement de ces impôts. Nous aurons l'occasion, monsieur le rapporteur général, monsieur le président de la commission des finances, de l'évoquer lors d'un projet de loi spécifique, qui sera présenté le 17 avril prochain en conseil des ministres et qui concernera la fiscalité locale.

des services sociaux. Nous nous attachons à simplifier pour les entreprises et les citoyens le recouvrement de l'impôt. Par ailleurs, la décrue du chômage sera accompagnée par le service public de l'emploi, renforcé notamment par la réforme de Pôle emploi. Nous assumons aussi que notre présence diplomatique soit redéployée en fonction de l'évolution des priorités stratégiques. Le Président de la République et le ministre des affaires étrangères ont eu l'occasion de l'évoquer. Voilà, madame la présidente, sans être plus long, quelles sont les grandes lignes de ce projet de budget. J'aurai l'occasion, pendant de longs débats, assisté d'Olivier Dussopt et Bruno Le Maire, de pouvoir répondre aux questions

L'an dernier, nous constations l'embellie économique dont vous bénéficiiez, messieurs les ministres, avec une apparente reprise solide de la croissance. Or, depuis le début de l'année, l'économie française croît deux fois moins vite que l'an passé.

la situation italienne. Je ne m'étends pas. En interne, il y a des incertitudes s'agissant de la consommation des ménages. En effet, le rebond attendu au troisième trimestre a été beaucoup moins fort qu'escompté, après la panne du premier semestre. Les ménages n'ont pas anticipé la fameuse augmentation du pouvoir d'achat que certains pouvaient attendre

Ces éléments sont d'autant plus importants que la sensibilité de la trajectoire budgétaire au scénario paraît importante, tandis que notre dette se rapproche dangereusement du seuil de 100 % du PIB.

mais j'y ajouterai le relâchement de l'effort de maîtrise de la dépense. J'y reviendrai. Vous vous êtes par ailleurs engagés dans des réformes qui ne sont pas financées, à l'instar de la suppression complète de la taxe d'habitation, mentionnée dans le programme de stabilité. Vous indiquez simplement qu'elle devra être financée par du déficit. Même en neutralisant la transformation du CICE, ce que vous avez indiqué à l'instant,

En tout état de cause, aussi peu ambitieux soit-il, le redressement des comptes publics prévu par le Gouvernement suppose la mise en oeuvre d'un programme de 14 milliards d'euros d'économies. Pour ce faire, malheureusement peu de réformes structurelles et un recours aux vieilles ficelles : des mesures de rabot sur les prestations sociales, déjà évoquées lors du PLFSS ; des « fusils budgétaires à un coup avec le décalage de certains allégements de charges sociales en octobre et le renforcement du cinquième acompte d'impôt sur les sociétés, qui vient ponctionner la trésorerie des entreprises ; des mesures structurelles d'ampleur très limitée et s'inscrivant assez largement dans la continuité du précédent budget. Ce sont, encore une fois, les secteurs du logement et de l'emploi qui produisent les efforts. Du côté de la sphère sociale, le Gouvernement se repose à la fois sur l'amélioration du contexte macroéconomique, s'agissant de l'assurance chômage, et sur les économies dégagées par les partenaires sociaux, pour les régimes complémentaires de santé S'il convient d'être prudent quant au respect de la trajectoire prévue pour la sphère locale, laquelle repose notamment sur un rebond des dépenses d'investissement et les effets de la contractualisation, les premières données d'exécution mettent en évidence la pleine détermination des collectivités locales à participer à l'effort de redressement des comptes publics. Au total, ce sont bien l'État et ses groupements qui porteront la totalité du besoin de financement, et ce pour la troisième année consécutive.

Du côté des recettes, la baisse de la fiscalité ne se matérialise pas vraiment. Sans le transfert aux administrations de sécurité sociale de 32 milliards d'euros, les recettes fiscales nettes de l'État seraient même en hausse de 18 milliards d'euros. On ne voit pas vraiment de baisse des prélèvements obligatoires.

n'ont pas accès à un mode de transport collectif. Même avec la prime à la conversion, l'achat d'un véhicule écologique reste trop coûteux pour nombre de Français. Par ailleurs, jusqu'aux annonces récentes du Président de la République, on constatait que les dispositifs de soutien que vous avez cités étaient en baisse.

la maîtrise des dépenses, nous restons sur notre faim. Alors que, sur le quinquennat, la loi de programmation des finances publiques prévoit une diminution de 1 % par an en volume, la cible pour 2019 s'avère d'ores et déjà dépassée, avec plus de 600 millions d'euros. Certes, la norme de dépenses « totales » devrait être respectée, mais il s'agit simplement d'une stabilisation. aussi de noter que certaines dépenses annoncées ne sont pas prises en compte dans le budget de 2019 ni dans la programmation pluriannuelle. Ainsi en est-il du service national universel : on ne sait pas si c'est 2 milliards ou 4 milliards d'euros de dépenses. Bizarrement, on n'en parle pas.

du champ d'intervention de l'État et des moyens qui lui sont assignés. C'est la raison pour laquelle la commission des finances proposera plusieurs amendements en seconde partie, afin notamment d'augmenter le temps de travail dans la fonction publique

vous savez très bien que les deux tiers correspondent en réalité à la compensation du manque à gagner lié à la hausse de la CSG intervenue l'an dernier. Surtout, bizarrement, vous oubliez les mesures de hausses de prélèvements décidées par les partenaires sociaux, qui vont peser sur les Français. Vous oubliez également, mais le Sénat y a remédié, le quasi-gel des allocations et des retraites. En réalité, faute de marges de manoeuvre budgétaires, votre politique revient, pour l'essentiel, à transférer du pouvoir d'achat d'une catégorie de ménages à une autre, et non à augmenter le pouvoir d'achat agrégé par une vraie action sur la croissance.

136 euros en 2018 et 538 euros en 2022 ! À partir de ces constats, la commission des finances proposera, comme elle l'a fait l'année dernière, de geler les tarifs de la TICPE à leur niveau de 2018, en supprimant la trajectoire prévue jusqu'en 2022. Nous ne ferons ainsi que confirmer le vote du Sénat l'an dernier.

Toujours sur le thème de la fiscalité écologique, la commission a également décidé d'instaurer une exemption de taxe générale sur les activités polluantes pour les déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets pour la part qui reste à ce jour non valorisable, c'est-à-dire environ 30 % des déchets.

du sujet de l'arbitrage des dividendes, mis en lumière par le journal et d'autres médias internationaux. Nous vous proposerons un dispositif qui permet d'éviter que des actionnaires non résidents de sociétés françaises échappent à la retenue à la source qui doit être appliquée sur les dividendes qu'ils perçoivent,

Madame la présidente, messieurs les ministres, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, nous entamons aujourd'hui l'examen en séance du projet de loi de finances pour 2019, après un long temps d'examen en commission. Je veux, en préambule, remercier l'ensemble de mes collègues de la commission des finances, mobilisés depuis depuis plusieurs semaines déjà pour étudier en détail les mesures budgétaires et fiscales de ce budget 2019. Près de cinq cents personnes ont d'ores et déjà été auditionnées par le rapporteur général et les rapporteurs spéciaux, et nous avons conduit plus de quarante heures d'auditions en commission plénière. J'associe à ces remerciements, bien sûr, l'ensemble de nos collègues des commissions saisies pour avis. Ces travaux préparatoires, qui sont d'ailleurs loin d'être terminés, nous permettront d'avoir des échanges nourris avec le Gouvernement. Ils témoignent de l'engagement Ils témoignent de l'engagement du Sénat à débattre et à amender ce projet de budget, qui, loin d'être un acte prévisionnel purement technique et comptable, ce qui justifierait que l'on en bâcle l'examen, constitue bien un acte fort et structurant de notre vie politique. J'en viens donc maintenant à l'analyse des principales mesures de ce projet de loi de finances. Pour ce qui concerne le cadrage macroéconomique, force est de constater que 2019 devrait marquer une déception, puisque la croissance s'établirait à 1,7 %, alors que le Gouvernement envisageait encore 1,9 % en juillet dernier. L'accélération de l'activité, dont certains prédisaient qu'elle résulterait quasi automatiquement- je n'ai pas dit magiquement -des réformes gouvernementales, ne s'est toujours pas manifestée et le contexte international est malheureusement de plus en plus incertain, comme vient de le rappeler l'OCDE. Dans le même temps, les efforts de redressement de nos finances publiques ne sont pas à proprement parler au rendez-vous. Je rappellerai simplement que, sous le précédent quinquennat, le déficit est passé de 5 % à 2,7 % du PIB, en diminuant chaque année, dans une conjoncture économique pourtant très défavorable. Entre 2017 et 2019, il passera de 2,7 % à 2,8 % du PIB. Nous ne faisons pas le minimum d'ajustement structurel requis par nos engagements européens nos résultats en matière de déficit public sont moins bons que ceux de nos principaux partenaires européens, et la dette publique continue de croître. Il y a lieu de nous en inquiéter dans un contexte de montée des incertitudes économiques dans le monde et dans la zone euro. J'en viens maintenant au volet fiscal de ce budget 2019, qui témoigne en creux non seulement de l'inefficacité, mais également de l'iniquité des mesures prises par la majorité gouvernementale l'an passé.

d'euros. J'ajoute que la baisse de la taxe d'habitation pour 7 milliards d'euros sur deux ans, si elle ne concerne pas les mêmes catégories de contribuables, n'en met pas moins à mal l'autonomie financière des collectivités locales. Faute de maîtrise réelle de la dépense publique, le Gouvernement n'a pu que compenser ces mesures fiscales coûteuses par la hausse d'autres impositions, dont les effets se prolongeront en 2019 : hausse de la CSG sur les retraités ou encore hausse graduelle, sur cinq ans, de la TICPE. À cet égard, le présent projet de loi de finances consolide le recours à la fiscalité énergétique, avec la suppression de l'exonération pour le gazole non routier, qui aura une incidence directe et très pénalisante sur nombre de petites et moyennes entreprises. Nombre d'orateurs reviendront sur ce point : la fiscalité énergétique sur les entreprises et les ménages progressera de 6,6 milliards d'euros sur deux ans, alors que les solutions alternatives n'existent pas encore, et donc ne permettent pas de réaliser la transition énergétique à laquelle nous aspirons tous. Le pouvoir d'achat d'un certain nombre de ménages modestes, en particulier retraités et ruraux, sera incontestablement amputé l'an prochain. Pour nombre de nos concitoyens, « budget du pouvoir d'achat » est bien loin de ses promesses. Sans doute y a-t-il là un puissant moteur de mécontentement, et il n'est pas nécessaire de chercher beaucoup plus avant les motifs de ce que nous constatons jour après jour sur nos routes et nos ronds-points. Pour ce qui concerne les dépenses, les mêmes missions que l'an passé sont sacrifiées, et en premier lieu les missions « Travail et emploi » et « Logement ». Comment dire mieux que ce sont les plus modestes des Français qui payent vos politiques ! Le Gouvernement fait le choix du désengagement du service public de l'emploi, alors même que le taux de chômage reste très élevé, au-dessus de 9 % de la population active il prend le risque de faire encore chuter la construction de logements sociaux, déjà amorcée, et il rabote les pensions et les prestations sociales en les désindexant. Ces orientations dessinent un désengagement des politiques sociales conduites par l'État, désengagement que le plan Pauvreté ne peut masquer. Le Gouvernement avait promis que, grâce au processus Action publique 2022, il trouverait les économies structurelles faisant aujourd'hui défaut. Il faut tout d'abord noter que, après avoir présenté comme un élément de crédibilité de la loi de programmation des finances publiques, il a refusé de rendre ses conclusions publiques. Notre commission, par mon intermédiaire, a dû menacer de recourir aux pouvoirs de la LOLF pour obtenir ce rapport. Or toute transformation de l'action publique doit se faire dans la transparence et le débat, surtout que le Premier ministre a affirmé, ici même, lors des questions d'actualité au Gouvernement, qu'il s'agissait d'un outil pour la réflexion du Gouvernement et qu'il a refusé de nous le transmettre. Bien sûr, la représentation nationale, elle, n'a pas à réfléchir Je note d'ailleurs à ce sujet que les parlementaires et les citoyens ne disposent toujours pas de l'ensemble des informations nécessaires pour pouvoir juger de la pertinence des mesures que le Gouvernement propose. L'an passé, dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances, j'avais présenté un amendement pour donner l'accès au « code source » des dispositions fiscales proposées par le Gouvernement, ce qui permettrait de ne pas dépendre, pour la moindre simulation fiscale, du bon vouloir de celui-ci et des services de Bercy. Cet amendement n'a pas été retenu par l'Assemblée nationale, mais je le présenterai de nouveau. Messieurs les ministres, nous sommes déterminés à refuser de légiférer à tâtons. Notre démocratie en sortirait d'autant plus renforcée.

Il a enrichi le projet de loi de lutte contre la fraude. Les membres du groupe de suivi que nous avons mis en place au sein de notre commission des finances proposeront, une fois de plus, une initiative transpartisane, pour soumettre les dividendes versés à des ressortissants étrangers à une retenue à la source effective. Il n'est en effet pas possible de demander à nos concitoyens des efforts s'ils n'ont pas le sentiment que tout le monde y consent et y concourt. J'espère ainsi que, malgré nos probables divergences sur un certain nombre de mesures contenues dans ce projet de loi de finances, nous saurons tous nous réunir autour de cette ambition. Nous passons à la discussion de la motion tendant à opposer la question préalable.

Madame la présidente, messieurs les ministres, mes chers collègues, loin de nous l'idée d'esquiver le débat avec le dépôt de cette question préalable. Ah ! Bien au contraire, nous voulons l'approfondir et lui consacrer plus de temps, faire en quelque sorte un point d'étape dix-huit mois après l'avènement du « nouveau monde ». Oh ! « Exaspération », cela peut paraître un mot assez fort, pour d'aucuns excessif, mais le fait est que c'est ce sentiment qui semble aujourd'hui profondément ressenti par un nombre important de nos compatriotes et concitoyens devant la politique menée par le Gouvernement. Les idées semblent d'ailleurs avoir pris de la vitesse pour se répandre dans l'opinion comme une traînée de poudre et nous sentons confusément que les choses ne peuvent continuer de la sorte. Il semble bien loin le temps du printemps 2017 où, après une victoire obligée, le Président de la République obtint la majorité parlementaire dont il avait besoin pour mener son programme. Cet argument des « engagements tenus », sans cesse ressassé depuis, commence tout de même à souffrir de n'avoir été partagé que par un peu plus de 15 % du corps électoral, soit la majorité la plus étroite obtenue par un vainqueur depuis l'inversion du calendrier électoral en 2002. Force est aujourd'hui de constater, depuis les rues de nos villes jusqu'aux péages d'autoroute en passant par l'entrée des usines ou le portail des écoles, que nous sommes à la recherche de ces fameux 15 %. Il faut dire que la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune, qui n'a nullement favorisé la relance de l'investissement productif, ne concernait que 350 000 ménages sur près de 40 millions de foyers fiscaux.

Le problème, c'est que cette fiscalité n'a souvent d'écologique que le nom ou le support et que son affectation est pour le moins sujette à caution. C'est vrai ! Je le sais pertinemment depuis que je participe aux travaux de cette assemblée, les recettes fiscales de l'État ont un caractère d'universalité qui ne souffre aucune contestation. Sauf que l'affectation demeure possible, dans des conditions précises, et que cela arrive notamment avec les taxes sur la consommation énergétique. Ainsi avons-nous un compte d'affectation spéciale « Transition énergétique » à l'intitulé séduisant et dont plus de 7 milliards d'euros de recettes, l'essentiel pour tout dire, est constitué d'un prélèvement de 39,75 % sur les recettes des taxes sur l'essence. Cela devrait réjouir quelques « gilets jaunes » ! Problème, voilà trois ans que ce compte d'affectation spéciale sert de « compte réservoir »- si je puis me permettre -, ce qui s'est traduit par le reversement cumulé de 1,8 milliard d'euros au budget général. La transition écologique s'est, une fois encore, inclinée devant les urgences de la petite cuisine budgétaire ! Chacun doit ici avoir en tête les données du problème. L'impôt sur les sociétés va rapporter, si tout va bien, environ 31,5 milliards d'euros en 2019, ce qui représente approximativement 1,3 % du PIB, pourcentage qu'on ne doit pas croiser très souvent chez nos partenaires européens. Cette réalité fait litière du faux débat mené pendant des années sur le taux de l'impôt sur les sociétés, qui a surtout besoin d'une sacrée réparation d'assiette pour que les PME à vocation locale, régionale ou même nationale n'aient pas l'impression de payer plus que les grands groupes familiarisés avec les prix de transfert, de transfert, le- pardonnez-moi l'anglicisme -la finance de l'ombre, le « double irlandais » ou le roboratif « sandwich hollandais ». De son côté, la TICPE, dont nous avons quelque peine à suivre les destinées maintenant qu'elle est affectée à des missions différentes, va dégager 37,7 milliards d'euros de recettes, hors taxes. Si on ajoute la TVA induite, on se retrouve avec une recette fiscale de 45 milliards d'euros, c'est-à-dire une fois et demie l'impôt sur les sociétés, qui connaît tout de même un certain nombre d'exceptions stupéfiantes. Certaines se comprennent, mais je dois dire que les plus récentes évolutions du tarif de la taxe posent question, notamment avec la fameuse contribution climat-énergie. Sous l'analyse de l'article 9 de la loi de finances initiale pour 2018, notre rapporteur général indiquait : « Eu égard au caractère Eu égard au caractère contraint de leur consommation énergétique et à leur faible capacité d'investissement en rénovation énergétique des logements ou en véhicules économes en énergie, les ménages ayant les revenus les plus faibles seront naturellement davantage impactés par une hausse de la fiscalité énergétique. C'est, du reste, la conclusion tirée par l'Observatoire français des conjonctures économiques, l'OFCE, dans une récente étude évaluant le programme présidentiel du Président de la République. L'OFCE a estimé l'impact selon les déciles de la composante carbone, en prenant pour hypothèse un prix de la tonne de carbone de 73 euros, soit un montant inférieur à la valeur de la tonne de carbone proposée par le Gouvernement pour 2021. Selon lui, l'impact selon les déciles de ménages varie d'un facteur 4 entre le premier- 1,8 % du revenu -et le dernier décile- 0,4 %. Les dépenses d'énergie de chauffage, considérées dans cette estimation comme incompressibles, contribuent fortement à ces disparités ». On peut effectivement décider de continuer sans se poser de questions, mais il est évident que nous irions alors au-devant de graves difficultés. Il y a de moins en moins de logique, mes chers collègues, à consacrer la TICPE à compenser aux collectivités locales, ce qui revient à leur faire payer une partie de la facture des fractures sociales, dans des conditions insatisfaisantes, le coût du revenu de solidarité active ou de la prise en charge de l'autonomie et de la dépendance. Là où nous devrions solliciter la sécurité sociale, la solidarité et la mutualisation, nous sommes en situation d'accabler de taxes l'automobiliste ou le locataire. La contribution climat-énergie n'est absolument pas consacrée à la moindre transition énergétique et son produit a, selon toute vraisemblance, alimenté quelques entreprises énergivores en allégements de cotisations sociales. Et demain, plus elle augmentera, plus elle servira à maintenir des milliers de salariés au SMIC, puisque ce niveau de rémunération est désormais libéré de toute contribution dite « patronale » au financement de la sécurité sociale. Nous avons pourtant bien d'autres choses à faire avec nos produits fiscaux, mais pas seulement. Dans un rapport qui vient de sortir sur le projet de loi d'orientation des mobilités, le Conseil économique, social et environnemental recommande d'utiliser de manière exclusive et fléchée le produit des taxes sur la consommation énergétique en faveur de la mobilité. Une telle idée ne nous semble pas dénuée d'un certain bon sens, même si elle nécessite de sérieuses adaptations de notre droit à la situation. Une démarche budgétaire plus audacieuse et plus en phase avec les attentes du temps aurait dû conduire à renoncer au transfert de 36 milliards d'euros de TVA vers la sécurité sociale pour compenser l'attrition de ses ressources et s'attaquer aux 17 milliards d'euros restants de la TICPE afin de renforcer les politiques de transition. N'en avons-nous pas besoin pour financer des plans climat-air-énergie territoriaux assortis d'objectifs précis en termes de réduction des déchets, de rationalisation de leur usage, d'investissement dans des véhicules non ou moins polluants ? N'en avons-nous pas besoin pour financer des plans de déplacements doux, des réseaux de transport collectif dignes de ce nom, évitant les effets de centralité, source de rupture de charges et de baisse de la qualité ? N'en avons-nous pas besoin pour promouvoir les circuits alimentaires courts, susceptibles de favoriser l'apprentissage du goût et de la qualité dès l'enfance, à l'école ? N'en avons-nous pas besoin pour promouvoir un renforcement des réseaux ferrés, même à vocation locale ou régionale, source d'un aménagement du territoire plus équilibré, permettant le moindre recours au transport automobile Aucun de ces enjeux, pas plus que les puissantes attentes sociales en matière d'emploi, d'action sociale, de logement, ne trouve grâce et place dans le projet de budget qui nous est soumis par le Gouvernement. Cet attachement aux choix opérés en 2017,

Je n'ai pas résisté au plaisir de lire l'objet de la motion : « Face aux attentes sociales et l'exaspération grandissante de la population devant la situation économique du pays, face aux enjeux fondamentaux que doit affronter notre pays, de par sa place en Europe et dans le monde, face aux questions de développement international équilibré, de transition énergétique et écologique, le projet de loi de finances 2019 n'apporte pas de réponses satisfaisantes, ni en termes de choix fiscaux, ni en matière d'affectation et d'utilisation de l'argent public. » Je suis tenté de dire

Le scrutin est ouvert.

C'est une maxime constante et reconnue dans tous les États du monde que les finances en sont la plus importante et la plus essentielle partie. C'est une manière qui entre en toutes les affaires, soit qu'elle regarde la subsistance de l'État en son dedans, soit qu'elle regarde son accroissement et sa puissance au dehors. Ces mots de Jean-Baptiste Colbert peuvent nous guider dans l'examen de ce projet de loi de finances. Ils doivent nous guider lors de nos débats, qui ne sauraient céder aux faiblesses susceptibles de surgir du besoin que nous aurions de nous faire des partisans en sacrifiant l'avenir au présent et les intérêts généraux aux requêtes particulières. L'intérêt général de la France, c'est celui de la prospérité de tous les Français et de tous les territoires. Tel était déjà l'objet central du projet de loi de finances pour 2018, il est encore le coeur de ce projet de loi Les premiers textes financiers du Gouvernement mettent aussi en lumière la constance et la clarté des choix. Et nous pouvons, je le crois, y adhérer : les Françaises et les Français, les salariés comme les entrepreneurs, ont besoin de la visibilité et de la stabilité qui ont pu manquer par le passé. Cela nécessite une trajectoire fiscale claire. Cette trajectoire est simple : elle passe par la baisse du taux de prélèvements obligatoires de un point et le financement des investissements productifs. Ces engagements sont concrets pour les Françaises et les Français, ainsi que pour les entreprises. S'agissant des ménages, les impôts baissent en 2019 de 6 milliards d'euros, principalement grâce à la suppression progressive de la taxe d'habitation et à la suppression des cotisations chômage et maladie. Nous sommes tous ici élus locaux, nous savons que la suppression de la taxe d'habitation représentera pour les Français, plus de 22 milliards d'euros de baisse d'impôts, dont l'évolution sera entièrement compensée par l'État pour les communes.

Il y a un choix, oui, celui d'alléger la fiscalité, avec des mesures fortes pour soutenir l'activité et l'emploi. La philosophie de notre groupe, La République En Marche, est assumée : elle vise l'inclusion de tous dans l'économie, car, la meilleure réponse à la pauvreté, c'est l'emploi. Nous voulons qu'en France le travail paie, qu'il permette d'accroître la production de richesses et qu'il finance, autrement que par l'impôt et par la dette, les protections que nous devons à tous nos compatriotes, en particulier aux plus fragiles. Je suis, comme vous tous, élu local. Les choix faits par le Gouvernement de clarté et de cohérence à destination des collectivités résonnent avec mon vécu. Cette année encore, la dotation globale de La dotation de soutien à l'investissement local, la DSIL, est maintenue à son niveau de 2017, soit 570 millions d'euros. Cette dotation est pérennisée par le Gouvernement,

Les collectivités ont une visibilité sur leurs recettes et l'assurance de pouvoir gérer leurs budgets. Après cinq années de coupes sans discrimination entre communes pauvres et communes riches, c'est une nouveauté bienvenue. Mes chers collègues, l'intérêt général de la France, c'est aussi changer notre modèle. Ce dernier repose sur la dépense publique financée par une dette qui frôle les 100 % du PIB. Le recul historique nous l'apprend avec clarté, quand il y a hausse des dépenses publiques, il y a hausse des impôts, hausse de la dette et baisse de la croissance. Ainsi, la période marque la plus grande baisse des dépenses publiques depuis cinq quinquennats : cette année, les dépenses publiques stagnent à 0 % en volume. Le déficit public pour 2019 est de 1,9 % du PIB, en retranchant la bascule du CICE

Conformément à la trajectoire votée par le Parlement, la dépense publique diminuera de trois points sur le quinquennat. Au regard des études économiques disponibles, ce rythme de consolidation budgétaire est le bon pour ne pas faire chuter la consommation privée et contraindre les ménages et les entreprises. En d'autres termes, nous arrivons à un moment où nous devons nous interroger sur des choix collectifs et budgétaires : malgré une dépense publique la plus élevée d'Europe, peut-on estimer que nos services publics sont les meilleurs ? Qu'en pensent les enseignants, les juges, les policiers et gendarmes ? L'État peut mieux faire, l'État doit mieux faire ! Mieux faire peut vouloir dire transformer les missions de l'État pour faire des économies, recentrer les actions, transformer le service public grâce au numérique. Mieux faire, c'est aussi répondre à l'enjeu de protection des Français. Le budget des armées connaît la plus forte augmentation de crédits depuis la guerre froide : l'effort pour nos armées sera porté à 2 % du PIB. C'était un engagement du Président de la République ; il est Protéger les Français signifie aussi renforcer nos forces de police et de gendarmerie. Cela commence par rattraper les 13 000 postes supprimés entre 2007 et 2012, mais cela signifie aussi repenser l'action de l'État pour la sécurité. Prendre conscience de la responsabilité qui nous incombe au moment de discuter le budget de la Nation, c'est aussi ne pas sacrifier l'avenir au présent. Nous pouvons nous imaginer Cyrus Smith, l'ingénieur né de l'esprit de Jules Verne, qui détourne un fleuve et maîtrise la nature, mais nous pouvons aussi imaginer, comme Simak, auteur de science-fiction, que, demain, l'Humanité ne sera qu'une légende dont parleront les chiens. Nous avons un grand devoir à l'égard des générations futures. futures. Nous autres parlementaires avons également deux choix : prétendre que la planète n'évoluera pas ou accompagner ce changement. Ces changements sont concrets, tangibles. Ainsi, dans l'un de ses scénarios sur le monde en 2040 récemment dévoilé, l'Agence internationale de l'énergie prévoit qu'un véhicule sur deux dans le monde sera électrique. Mes chers collègues, la la sagesse du Sénat doit être au service de l'intérêt général et de la Nation. Notre groupe sera, en conséquence, attentif sur les propositions qui pourraient sacrifier l'avenir, qu'il s'agisse d'aggraver le déficit public par des mesures sectorielles, de flatter ou satisfaire l'ego de quelques secteurs au détriment de tous les Français qui devront payer, ... Ils paient déjà ! ... qu'il s'agisse, par exemple, de faire croire aux Français que l'environnement n'est pas un sujet,

Madame la présidente, messieurs les ministres, mes chers collègues, selon les simulations menées à l'aide du modèle Ines, le revenu disponible moyen par ménage, en euros constants, serait, en 2016, inférieur de 1,2 % à son niveau de 2008. Les réformes fiscales visant le redressement structurel des comptes publics engagé à la suite de la crise économique, la hausse du chômage et du temps partiel et les évolutions démocratiques sont sûrement des facteurs qui peuvent expliquer cette diminution. Sans les réformes fiscales intervenues entre 2008 et 2016, le revenu disponible moyen des ménages aurait été supérieur de 1,4 % en 2016. Les effets de ces réformes diffèrent selon la place des ménages dans la distribution des niveaux de vie. Les ménages les plus aisés- mais c'est bien le minimum -ont été les plus mis à contribution les 5 % du haut de la distribution ont vu leur revenu disponible annuel diminuer de 5 640 euros sous l'effet des mesures nouvelles concernant les prélèvements- hausse des cotisations sociales, création d'une tranche d'impôt sur le revenu à 45 %, imposition au barème de l'impôt sur le revenu des revenus du capital, etc. Les ménages les plus modestes ont bénéficié de la politique sociale et des amortisseurs sociaux encore existants : les 5 % les plus modestes ont vu leur revenu disponible annuel s'accroître de plus de 450 euros et les 5 % de la tranche au-dessus l'ont vu s'accroître de 890 euros du fait des réformes des prestations- revalorisation des minima sociaux, création de la prime d'activité, etc. Messieurs les ministres, les réformes des prestations et prélèvements mises en oeuvre en 2017 ont, à nos yeux, un impact quasi nul sur les inégalités de niveau de vie. Ce que je viens de citer ici, mes chers collègues, ne pouvait figurer dans le document de présentation du budget pour 2019, puisque ces lignes sont issues d'une fort instructive note d'actualité de l'INSEE, publiée avant-hier. Si elle ne loin de là ! -les politiques du précédent quinquennat, elle témoigne, en revanche, que les quelques garde-fous encore préservés pour freiner l'aggravation des inégalités sociales ont sauté en 2017, avec ce que nous appelons l'avènement d'une course folle vers un ultralibéralisme sans limites. Oui, c'est bien un nouveau projet de société qui est à l'oeuvre, encore plus violent pour les salariés, pour les familles populaires et les classes moyennes, un projet toujours plus protecteur pour les actionnaires des grandes entreprises et pour les marchés financiers. Ainsi, si l'on compare la première année du précédent quinquennat, largement rejeté par les milieux populaires, et la première année du quinquennat en cours, c'est-à-dire les lois de finances initiales pour 2013 il semble bien que quelques données ont évolué et qu'elles n'ont certainement pas contribué à améliorer la situation de la grande majorité de nos compatriotes. Dans la loi de finances pour 2013, on avait ainsi prévu, entre autres, de percevoir les recettes suivantes l'impôt sur le revenu, 72,8 milliards d'euros ; pour l'impôt sur les sociétés, 52,3 milliards d'euros, malgré le CICE ; pour la TVA, 141,8 milliards d'euros TICPE, 13,8 milliards d'euros. Et nous avions une prévision de 85,2 milliards d'euros en remboursements et dégrèvements d'impôts d'État et de 10,9 milliards d'euros pour les impositions locales. Devenu sénateur et rapporteur de la mission « Remboursements et dégrèvements je me devais de le souligner. La part de la fiscalité indirecte était déjà importante dans l'ensemble des recettes, mais il n'en demeure pas moins que la situation n'était pas celle d'aujourd'hui. Dans le projet de loi de finances

par le transfert de plus de 36 milliards euros pour compenser les allégements sociaux ; pour la TICPE, 17 milliards d'euros. Par ailleurs, le montant des remboursements et dégrèvements continue son ascension.

17,5 milliards vers les ménages et environ 13,5 milliards vers les collectivités locales. Quand on regarde l'évolution des recettes fiscales, on constate l'effondrement du produit de l'impôt sur les sociétés, celui-ci se situant à environ 1,3 % du produit intérieur brut. Pour dire les choses simplement, cela représente quatre jours et demi de production, c'est-à-dire de travail des salariés. C'est un peu comme si les entreprises de notre pays commençaient l'année 2019 en se disant que, dès le 6 janvier, elles auraient fini de payer l'impôt sur les sociétés

Les ménages salariés, retraités et autres de notre pays vont donc, mes chers collègues, laisser 60 milliards à 65 milliards d'euros en 2019 en ristourne aux actionnaires des entreprises. C'est l'équivalent d'un impôt invisible

où les bases d'imposition vont, contre toute logique économique, s'éloigner de la sphère de la production pour se concentrer sur les revenus, inégalitaires, et la consommation sous toutes ses formes. En lieu et place d'un impôt sur le revenu plus progressif, comme nous le demandons, avec une augmentation du nombre de tranches et une modification des taux, nous aurons, demain, un impôt sur le revenu rendu moins progressif par le traitement de faveur accordé aux revenus du capital et du patrimoine, dont la CSG, transformée en impôt de base, sera l'élément le plus dynamique.

est, nous aurons, à n'en pas douter, de nouveaux droits de consommation sur les alcools, le tabac, les boissons gazeuses, les boissons avec édulcorants, la consommation en général, l'utilisation de l'air, le recours à l'énergie et aux carburants, etc. Voilà cinq ans, évoquant ici même notre opposition à la mise en place de la contribution climat-énergie, soulignait : « Derrière l'article 20 se cache un nouvel alourdissement de la fiscalité indirecte pour les ménages à hauteur de 230 millions d'euros dès 2014, et de 2,7 milliards d'euros en 2016. « Le prix du plein Le prix du plein d'essence ou de gazole, la facture de chauffage au gaz ou au fioul vont augmenter sans que les intéressés puissent y faire grand-chose. La grande remise à plat de notre système fiscal ne pourra ignorer la situation des familles contraintes d'utiliser leur véhicule personnel pour aller travailler ou dont les logements collectifs sont chauffés grâce au fioul ou au gaz. « L'article 20 nous éclaire sur le sens de certaines réformes fiscales : avant deux ans, compte tenu de la montée en charge de sa composante carbone et des pleins effets du crédit d'impôt pour la compétitivité et pour l'emploi, la TICPE va se transformer en recette fiscale plus importante que l'impôt sur les sociétés. Une telle logique nous déroute quelque peu. « En effet, le produit de cette hausse sera affecté non pas à la transition écologique, mais à la réduction des cotisations sociales des entreprises dans le cadre du trop fameux CICE. Les rôles sont donc clairement partagés : d'un côté, les entreprises collectent l'impôt et le facturent en dernier ressort au consommateur avant de percevoir le produit du CICE, de l'autre, les consommateurs ont le droit de payer le tout directement ou indirectement, sans espérer autre chose qu'un hypothétique mouvement d'embauche dans le secteur privé. Nous ne pouvons évidemment que proposer la suppression de cet article, qui pervertit totalement le bien-fondé de la fiscalité écologique et témoigne, une fois encore, du fait que l'approche fiscale des problèmes environnementaux n'est pas la bonne. » Ces propos ont été Si j'ai jugé utile ce rappel, c'est que nous sommes en des temps où les amalgames faciles nourrissent l'antiparlementarisme le plus éculé ... Ah ! ... et brouillent l'écoute que nous devrions avoir à l'égard des attentes de nos compatriotes. Enfer fiscal pour le plus grand nombre : voilà ce que devient notre pays avec ce projet de budget ! Et je ne dis rien des dépenses dans le détail. Pour ne citer qu'un exemple, on rappellera que l'on se félicite de l'adoption du prélèvement à la source, car il permettra de réaliser 1,4 milliard d'euros d'économies sur les aides personnelles au logement ! Cela n'a rien à voir ! Quel bonheur que de risquer de perdre l'anonymat sur ses revenus auprès de son employeur pour être sûr de ne plus toucher d'allocations logement ! Mais l'enfer doit bien avoir un paradis. l'enfer doit bien avoir un paradis. Oui, la France est en train de devenir un paradis, un paradis financier. En effet, 31,5 milliards d'euros d'impôt sur les sociétés et un peu moins de 30 milliards d'euros de fiscalité locale pèsent-ils beaucoup au regard des 100 milliards d'euros de remboursements et dégrèvements accordés aux entreprises, s'ajoutent les allégements de cotisations sociales, largement majorés cette année par l'intégration du CICE et les mesures retracées dans l'évaluation des voies et moyens, comme les 34 milliards d'euros du régime des groupes ou les 7 milliards d'euros de la « niche Copé » ? Nous ne sommes plus très loin de ressembler à un paradis financier un paradis financier pour actionnaires et individus fortunés, privés d'impôt de solidarité sur la fortune, dotés d'un prélèvement forfaitaire et bientôt pourvus d'une exemption inégalée de leurs donations.

qu'elle aggrave les ressentiments déjà profonds dans notre société, ce que nous devons absolument éviter. C'est cette situation que nous allons résolument combattre avec nos amendements, pour montrer qu'une autre voie est possible face à cette politique, dont plus personne ne pourra maintenant nier qu'elle est ultralibérale, et donc ultralibérale. Nous ne le ferons pas pour alimenter l'idée que l'impôt est par nature un enfer.

Madame la présidente, messieurs les ministres, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, pour le Gouvernement et le Parlement, la présentation et le vote d'un budget constituent l'acte majeur de l'année, celui qui sous-tend toute la politique gouvernementale et dessine les frontières des majorités et des oppositions. Comme les années précédentes, il convient de replacer l'examen du projet de loi de finances dans un contexte historique, économique, social et financier, à l'échelon tant national qu'international. L'environnement international n'a jamais été aussi perturbé et incertain, avec des foyers de conflit au Moyen-Orient, une politique isolationniste des États-Unis, une volonté expansionniste de la Chine et un manque évident de cohésion en Europe. Sur le plan économique, on assiste à une complexification des échanges internationaux, à une plus grande volatilité des cours du pétrole et des matières premières, à un tassement des perspectives de croissance en Europe ainsi qu'à la persistance de nos faiblesses structurelles dans le secteur industriel. Le contexte historique national, c'est en fait l'état des lieux dégradé de la maison France au début de ce quinquennat en termes de dette, de déficit public, de balance commerciale et de niveau de chômage. Les gouvernements précédents, malgré des efforts parfois méritoires, n'ont pas réussi à inverser les tendances négatives de ces indicateurs. C'est le défi que le Gouvernement doit relever : réussir là où ses prédécesseurs ont échoué. Ce constat devrait conduire ceux qui ont gouverné ou soutenu les politiques publiques lors de la dernière décennie à la plus grande modestie ainsi qu'à plus de réserve dans leurs critiques et leurs propositions, mais aussi le Gouvernement à respecter une certaine prudence dans l'affirmation de ses certitudes. de loi de finances pour 2019 est à la fois un budget de transformation et de transition. En effet, si le déficit budgétaire atteint 98,7 milliards d'euros, il aurait été à périmètre comparable à 76,3 milliards, soit inférieur de 3,7 milliards d'euros d'euros au déficit prévu pour 2018. Cet écart de 22,4 milliards d'euros s'explique par le basculement du CICE en diminution de cotisations sociales pour les entreprises,

mais aussi le décalage d'un mois de recettes d'impôt sur le revenu lié à la mise en place du prélèvement à la source, mesure légèrement compensée par l'avènement d'un cinquième acompte d'impôt sur les sociétés pour les entreprises. Ce projet de loi de finances nous inspire un certain nombre de satisfactions, mais aussi quelques réserves, interrogations et inquiétudes. Au rang des satisfactions figurent : le respect de la trajectoire budgétaire fixée dans la loi de programmation financière pour les années 2018 à 2022, avec un déficit public de 1,9 % du PIB majoré à 2,8 % du fait de dispositions exceptionnelles- je pense au CICE ; la construction budgétaire fondée sur des hypothèses macroéconomiques jugées crédibles par la Cour des comptes, laquelle estime raisonnable le maintien d'un taux de croissance à 1,7 % du PIB un maintien pour la deuxième année consécutive des concours financiers aux collectivités territoriales, avec une enveloppe normée stabilisée à 40 milliards d'euros ; une augmentation du pouvoir d'achat estimée par le Gouvernement à 6 milliards d'euros, inflation et fiscalité écologique incluses, mais qu'il faut ramener en progression nette aux environs de 3 milliards d'euros, pour tenir compte du plafonnement de l'évolution des retraites et pensions enfin, une légère baisse du niveau des prélèvements obligatoires, qui devrait s'établir à 44,2 % en 2019, au lieu de 45 % en 2018. Des réserves et interrogations que l'on peut formuler,

Si la hausse et la variation du prix des carburants sont bien principalement imputables à l'évolution du prix du pétrole brut, le manque de clarté dans le fléchage du produit de cette taxe a handicapé la pédagogie du Gouvernement et n'est pas étranger à la grogne de nos concitoyens. La seconde réserve- peut-être plus personnelle -porte sur la désocialisation des heures supplémentaires, qui est bien l'introduction de 600 millions d'euros en 2019 et de 2 milliards d'euros en année pleine de pouvoir d'achat pour les salariés accomplissant des heures supplémentaires. Cette mesure, certes populaire, représente malgré tout un effet d'aubaine, qui a quelques inconvénients et effets pervers, en ne concernant qu'à peine la moitié des salariés du secteur privé, en annulant la création de 12 000 emplois par an et en n'ayant aucun effet de levier sur la croissance et la compétitivité J'en viens aux inquiétudes et tiens à rappeler la gravité que représente un déficit budgétaire, même ramené à 76 milliards d'euros. Il faudrait en effet, par exemple, doubler les recettes de l'impôt sur le revenu pour retrouver l'équilibre budgétaire. Par ailleurs, la dette continue de progresser, avec une charge annuelle de 42,5 milliards d'euros. La dépense publique ne baisse pas et la diminution des emplois dans les services de l'État est assez faible, de l'ordre de 4 000 en 2019, ce qui reporte à la deuxième moitié du quinquennat tout l'effort auquel le Président de la République s'était engagé. Une autre crainte porte sur les choix qui pourraient être faits par nos compatriotes entre la consommation, l'investissement et l'épargne. Les Français sont déjà parmi les plus gros épargnants du monde, avec 5 100 milliards d'euros de patrimoine financier hors immobilier des ménages. Si les gains de pouvoir d'achat s'orientent vers le renforcement d'une épargne défensive, épargne de précaution peu risquée et peu rémunératrice, cela pénalisera lourdement l'investissement et la consommation des ménages, de même que le renforcement des capitaux propres des entreprises. Ainsi, la hausse de 0,7 % de pouvoir d'achat du deuxième trimestre de 2018 a pris intégralement le chemin de l'épargne, dont les flux collectés sont passés sur cette période les ministres, les ressorts d'une reprise économique en 2019 sont bien présents sur le plan technique et financier, mais ils risquent d'être neutralisés par une approche psychologique de la situation assez pessimiste de la part de nos compatriotes, largement amplifiée par les événements et effets médiatiques. En conclusion, je dirai que notre appréciation de ce projet de budget est plutôt contrastée, même si elle demeure globalement positive. Le groupe du RDSE ne remet pas en cause l'orientation générale de de la politique du Gouvernement et des importantes réformes structurelles qui sont ou seront engagées. Nos propositions par voie d'amendements concerneront des ajustements mineurs destinés à mieux répondre à certaines situations, sans effets significatifs en termes de masse financière. Dans la ligne directrice qu'il s'est fixée, l'exécutif doit poursuivre les réformes engagées, accentuer ses efforts pour diminuer la dépense publique et le niveau des prélèvements obligatoires. La majorité du groupe du RDSE ne s'associera pas aux amendements qui pourraient infléchir de manière trop grossière ce projet

un budget ne peut être bon que s'il est, également, au service d'une bonne politique. J'ai observé avec intérêt les premiers pas de ce gouvernement et j'ai approuvé les mesures qui avaient trait à la simplification et à la relance de l'économie et de l'investissement. Force est de constater aujourd'hui que nous sommes loin d'une bonne politique, dans la mesure où certains vieux démons de Bercy ont repris le dessus. Un exemple emblématique en est, à mes yeux, la suppression de la taxe d'habitation. Plus que la volonté de tenir une promesse, il est question pour Bercy de satisfaire un vieux rêve, à savoir remplacer l'autonomie fiscale et financière des collectivités territoriales par des dotations. Nous serions dans la main de Bercy. Or cette décision est tout à la fois absurde et injuste. est absurde, car elle conforte ceux des élus locaux qui avaient voté les impôts les plus élevés et condamne ceux qui, dans un souci de bonne gestion, avaient voté de faibles impôts et n'auront aucune solution pour dégager des marges de manoeuvre en cas de besoin. Cette décision est injuste, dans la mesure où elle donne le plus de pouvoir d'achat à ceux qui ont déjà les revenus les plus élevés. Je rappelle que 30 % de nos

On nous présente des moyennes départementales, mais on ne nous dit rien de la fourchette. Combien de pouvoir d'achat en plus pour ceux qui habitent dans des hôtels particuliers ? Il aurait été plus juste de proposer un abattement forfaitaire pour tous. Cette décision grève le budget de l'État sans provoquer en retour de création de richesses. Elle oblige le Gouvernement à faire la course aux recettes nouvelles, d'où l'explosion des taxes et prélèvements.

Le doublement de la prime pour changer de véhicule ne résoudra rien. Ceux qui n'ont pas les moyens financiers ou ceux qui viennent de s'engager en souscrivant un crédit ne profiteront pas de ces dispositions nouvelles.

Une bonne politique aurait consisté à consacrer l'argent des taxes à construire des infrastructures, facilitant les alternatives. Combien y a-t-il de postes de recharge à hydrogène en Allemagne ? Combien en compte-t-on en France ? Combien de postes pour les véhicules au gaz ? Combien pour ceux qui vont rouler au E100 ? On n'a pas consacré l'argent des taxes à permettre aux gens de faire d'autres choix. Devant le ras-le-bol exprimé par nos concitoyens, on a l'impression d'un affolement général, donc d'un accroissement de la complexité, d'un éloignement des centres de décision, d'une volonté de la technocratie de vouloir faire le bonheur des citoyens et des collectivités à leur place, souvent contre eux. Un bon budget technique n'est pas nécessairement un bon budget politique. Il faut le regretter, car notre pays a des défis énormes à relever. Rien n'est dit ou fait pour corriger le déficit de notre commerce extérieur. Pourtant, il n'est pas neutre par rapport à notre déficit public, qui atteindra les 100 milliards d'euros, et à notre endettement, qui atteindra 1 000 milliards d'euros. Il serait temps de se consacrer à l'essentiel, l'accroissement de la création de richesses.

L'enfant de ce couple, c'est un État obèse, écrasant l'activité économique par sa gloutonnerie fiscale. Cette situation fait de la France le dernier de la cordée européenne. Pour preuve, depuis une semaine, nous vivons à crédit. Eh oui ! Pendant quarante-six jours en effet, les services de l'État sont payés à crédit. Seules la Pologne et la Roumanie font moins bien que nous. Le résultat, c'est un déficit très élevé : 100 milliards d'euros avec le CICE, 80 milliards d'euros sans le CICE, soit à peu près 30 milliards d'euros de plus qu'en 2017.

Certains diront que, depuis quarante ans, on a tout essayé pour rétablir les comptes publics. Il n'en est rien. On a tout essayé, sauf la baisse de la dépense publique. Maîtriser la dépense ne suffit pas. La réduire est une nécessité. Il ne suffit pas de le dire, messieurs les ministres. Il faut le faire. Les discours, c'est bien ; les actes, c'est mieux. Que proposez-vous ? Vous verrez au cours du débat ce que nous proposerons, monsieur le ministre, et j'espère que vous approuverez nos dispositions d'économie.

Pour les seules dépenses de l'État, en 2019, ce sont 6 milliards d'euros de plus que vous nous proposez, messieurs les ministres. Sur trente missions, vingt sont à la hausse et seulement dix à la baisse.

que le pouvoir d'achat moyen des Français avait baissé de 440 euros par an entre 2008 et 2016, notamment du fait du choc fiscal du quinquennat Hollande.

Personne n'est dupe de cette tromperie, qui a légitimement causé la colère de millions de Français, « gilets jaunes » ou pas. Alors, si l'on ne doit retenir qu'une seule chose dans nos discussions budgétaires, c'est que les dépenses d'aujourd'hui sont les impôts de demain. Résultat, on a dépassé les 1 000 milliards d'euros d'impôts et de taxes collectés dans notre pays. La France bat cette année deux records : le niveau des dépenses publiques- elle est le premier pays de l'OCDE -et celui des impôts et taxes- elle est le premier pays de l'Union européenne.

jusqu'au 27 juillet, on travaille pour l'État et toutes les caisses de sécurité sociale et de retraite ; à partir du 27 juillet, on travaille pour soi-même. Messieurs les ministres, au vu de ce projet de budget, je crains que la France ne cesse de sitôt d'être le pays le plus dépensier, donc le plus taxé. plus dépensier, donc le plus taxé. Pour moi, un bon gestionnaire de l'argent public devrait être sincère, prudent et économe. Messieurs les ministres, votre gouvernement est-il sincère ? Oui, sans aucun doute, et c'est un gros progrès. Est-il prudent ? Un peu, mais il peut à mon avis mieux faire en la matière. Économe ? Assurément pas. Il est urgent de progresser dans cette direction,

prises pour son application, la commission de la culture, de l'éducation et de la communication a émis un avis favorable- 12 voix pour, 1 voix contre -à la nomination de M. Gilles Bloch aux fonctions de président de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.